Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les dispositifs de soutien aux entreprises inclus dans la mission « Économie » sont tellement hétérogènes que les gouvernements successifs semblaient s'être résolus, année après année, à une simple logique de rabot.

super-rabot » n'est pas forcément une critique, car il est nécessaire de mettre de l'ordre parmi les multiples aides directes ou indirectes, prêts, garanties, actions collectives de formation, de promotion ou encore de mutualisation- sans même parler des crédits d'impôt et autres dépenses fiscales. leur accumulation progressive, leur sédimentation et leur gestion en silos avaient fini par les rendre illisibles et impropres à incarner les priorités politiques d'un gouvernement, quel qu'il soit. Une partie de la baisse des crédits s'explique aussi par la suppression de la dotation de 40 millions d'euros à Bpifrance Garantie. Non que l'État se désengage, mais Bpifrance dispose, au moins pour l'instant, de la trésorerie nécessaire pour assurer cette mission. Je me félicite toutefois qu'une ligne de crédits, certes symbolique- 10 000 euros -, ait été rétablie par l'Assemblée nationale, sur l'initiative d'Olivia Grégoire, pour préserver le lien entre le Parlement et Bpifrance.

Ce que nous percevons entre les lignes, c'est un désengagement progressif et délibéré de l'État, comme une manière de dire aux collectivités territoriales, et d'abord aux communes et aux régions : c'est maintenant votre travail Or les choses ne sont pas aussi simples. Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales, le maintien de dispositifs ponctuels, au demeurant très modestes, constitue une forme de soutien complémentaire : pour ainsi dire, un « plan B », lorsqu'il n'existe pas de « plan A » au niveau local. Ce n'est pas grand-chose pour l'État, mais c'est beaucoup pour les territoires.

La même remarque vaut pour les chambres de commerce et d'industrie. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler lors de l'examen de la première partie, alors que la revue de leurs missions se poursuit et que les mesures d'accompagnement du projet de loi PACTE ne sont pas encore votées, les CCI font face à une nouvelle baisse de leur

Madame la secrétaire d'État, toutes les autorisations d'engagement ont aujourd'hui été consommées, et seuls des crédits de paiement seront débloqués en 2019. Or il est aujourd'hui clair que les sommes prévues ne suffiront pas. Elles ne suffiront pas, d'abord, à résoudre les problèmes que nous constatons tous dans nos territoires. Seuls 10 % des locaux situés dans la zone d'initiative publique sont, à ce jour, éligibles à la fibre optique, contre 56 % des locaux de la zone d'initiative privée, plus dense, donc plus rentable. La possibilité de demander des engagements contraignants aux opérateurs, les fameux appels à manifestation d'engagements locaux, ou ne résoudra pas tous les problèmes. L'ouverture d'un guichet de cohésion numérique pour financer des technologies alternatives- 4G fixe et satellite -dans les zones reculées va dans le bon sens, mais ce guichet ne représente que 100 millions sous forme de subventions individuelles de 150 euros par équipement, sans engagement des opérateurs à maintenir un tarif attractif au-delà d'un certain délai. Surtout, si les crédits actuels permettent de financer la couverture du territoire à 100 % en très haut débit, ce qui compte, à terme, c'est bien l'objectif d'une couverture à 100 % en fibre optique. Il faut dès aujourd'hui se poser la question de l'après-2022. Je ne parle pas seulement du déploiement des réseaux, mais aussi de leur maintenance à long terme. Demain, plusieurs réseaux coexisteront en France, ce qui constituera une rupture avec l'époque du monopole d'Orange sur le réseau cuivre. C'est un défi majeur. Le ministre chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie, a confirmé que l'État continuerait à accompagner les collectivités territoriales les crédits du Grand Plan d'investissement. On évoque un montant total de 700 millions d'euros, dont 200 millions dès 2020.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil national de l'industrie, réuni par le Premier ministre le 22 novembre dernier, s'est ouvert sur une excellente nouvelle

c'est une vérité que nous devons tous partager ! Pourtant, madame la secrétaire d'État, la situation de notre commerce extérieur reste alarmante : l'année dernière,

125 000 entreprises exportatrices en France, contre 360 000 en Allemagne et 200 000 en Italie. Mais, heureusement, les choses changent. Comme vous le savez, depuis 2015, Business France rassemble au sein d'une même agence les missions d'accompagnement à l'export et de promotion des investissements étrangers en France. Principal opérateur rattaché à la mission « Économie », Business France n'a pas à rougir de son bilan : ses objectifs pour la période 2015-2017 ont tous été atteints, et avec des crédits budgétaires en baisse.

Reste que l'efficacité de cette politique publique était jusqu'à présent entravée par l'éclatement des acteurs et la superposition des compétences. Le coeur du problème réside paradoxalement en France, dans ces territoires d'industrie dont j'ai parlé il y a quelques instants. Jusqu'ici, Business France n'avait pas de présence opérationnelle sur le territoire, territoire, mais seulement à l'international. Or, avec une volonté affirmée de se réinsérer dans nos territoires, Business France a la possibilité, avec ses 100 conseillers

Contrairement à la première tentative, en 2015, les choses ont l'air de très bien se passer. Tout en apportant notre soutien enthousiaste à cette réforme, nous pensons, madame la secrétaire d'État, qu'il faut aller encore plus loin. C'est le sens de la proposition que nous avons soumise à la commission des finances, qui l'a retenue

Tout en devenant familier des métiers et du savoir-faire de l'entreprise, cet étudiant ou ce jeune diplômé resterait tout entier mobilisé pour sa mission de projection à l'international. Il assurerait le lien avec la « Team France Export » la plateforme des solutions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a observé avec inquiétude la forte baisse des crédits d'interventions en faveur des entreprises du programme 134 de la mission « Économie », d'autant qu'il est concomitant du désengagement forcé d'autres acteurs de l'accompagnement des entreprises, les chambres de commerce et d'industrie. Dans ce cadre, elle a porté son attention sur trois sujets particuliers. Le premier est la disparition annoncée du FISAC. Alors que le Gouvernement clame sa volonté de redynamiser les centres-villes, il fait disparaître ce fonds destiné au maintien des commerces de proximité, notamment en milieu rural. Or l'enjeu de revitalisation commerciale ne concerne pas seulement les 222 lauréats du plan « Action coeur de ville ». Il est donc impensable de supprimer totalement le FISAC, même si on l'étouffe à petit feu depuis cinq ans.

du fait de la montée en puissance de la compétence économique des régions et du rôle joué par les opérateurs spécialisés de l'État, Bpifrance et Business France. Toutefois, il importe que cette évolution n'aboutisse pas à l'abandon pur et simple par l'État de toute action micro-économique. Il faut au Il faut au contraire un recentrage fondé sur les principes de subsidiarité et de garantie des équilibres économiques nationaux, car l'État est le seul à même d'avoir une vision du développement économique qui dépasse l'échelle régionale. L'État déconcentré doit jouer le rôle de coordinateur des acteurs publics et parapublics dans la mise en oeuvre d'une stratégie d'équilibre économique des territoires, en favorisant les synergies entre acteurs. Il faut également conserver des capacités d'intervention ponctuelle ciblée, complémentaires de celles des autres acteurs. Le troisième sujet sur lequel nous entendons insister est l'organisation des acteurs du monde consumériste. le projet de loi de finances poursuit la réduction des crédits d'intervention en faveur des acteurs du monde de la consommation, la modicité et la réduction constante des moyens financiers mis en oeuvre par l'État en en faveur de la protection du consommateur doivent incontestablement conduire à une réflexion d'ensemble sur l'architecture du système de protection des consommateurs. Or, plutôt que de s'engager dans cette voie, le Gouvernement mène malheureusement une politique de rabot continue, qui paralyse progressivement l'action des acteurs sans les engager dans un modèle d'organisation alternatif. La commission a donc décidé de se saisir de cette question et de réfléchir au positionnement des différents acteurs pour proposer des pistes d'évolution.

Sous réserve de l'adoption de ses deux amendements, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ma contribution portera sur le volet numérique et postal. En ce qui concerne la mission de transport de presse par La Poste, il conviendrait, à l'avenir, d'associer davantage les représentants du secteur de la presse à la définition

Sur cette question des ondes, il me semble également qu'un travail renforcé de pédagogie auprès du grand public s'impose, afin que chacun soit en mesure d'apprécier correctement les risques et connaisse mieux les bonnes pratiques. du plan France Très haut débit, il est nécessaire d'amplifier l'accélération en cours dans les zones moins denses pour atteindre le rythme de 4 millions de prises par an. Le Gouvernement devra également définir d'ores et déjà les nouvelles orientations de l'après-2022, afin d'offrir une meilleure lisibilité aux acteurs et investisseurs. qui est du guichet de cohésion numérique, il conviendra de s'assurer de la bonne articulation entre les aides octroyées par ce guichet et celles versées par les collectivités territoriales afin de développer les technologies alternatives à la fibre, notamment l'Internet par satellite. sur les entreprises de réseau, ou IFER, pour les nouveaux déploiements opérés dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, même si celle-ci est rédigée. Une réflexion sur la fiscalité applicable aux opérateurs de communications électroniques

et le transfert de son personnel à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Seul le pôle restera à Bercy. Globalement, l'Agence du numérique a su mener à bien des missions diverses et particulièrement évolutives. de l'inclusion numérique ne dispose toutefois pas des moyens de ses ambitions, même en prenant en compte les dernières mesures rendues publiques en septembre dernier. Il s'agit pourtant d'un enjeu majeur, qui concerne 14 millions de nos concitoyens, soit 28 % de la population. devra mener à bien la mise en oeuvre du plan France Très haut débit et du plan pour l'inclusion numérique. La plus-value à attendre de cette absorption reste encore à démontrer, car l'ANCT devra être aussi agile et souple que le fut l'Agence du numérique. L'enjeu est d'éviter les pertes d'expérience

industrielles restent fragilisées et que la balance commerciale française est largement déficitaire, les moyens de la mission « Économie » se détournent peu à peu de l'industrie. Mes chers collègues, le symbole est fort : la ligne Action en faveur des entreprises industrielles est tout simplement supprimée Ses crédits sont absorbés par une nouvelle action, Industrie et services, dont le champ très large complique grandement le travail de contrôle budgétaire du Parlement. Certes, les crédits de paiement de la mission sont en légère hausse, mais les autorisations d'engagement chutent de 17 %. comment l'État entend-il s'engager dans une politique industrielle de long terme aux côtés de nos entreprises ? Moins d'un euro sur trois de la mission « Économie » est désormais alloué à des dépenses d'intervention

qu'elles deviennent un acteur de plus en plus important du développement économique. Tout de même, nous ne devons pas mettre un terme brutal au soutien de l'État ! La commission des affaires économiques a donc déposé un amendement à maintenir le niveau actuel de dotation globale pour les actions de soutien à la compétitivité des entreprises : 3,2 millions d'euros de dotation seront ainsi préservés. Alors que les taxes pèsent toujours plus sur les entreprises industrielles, avec la double peine de la fiscalité énergétique et de la fiscalité de production, le Gouvernement entend, de surcroît, étrangler le financement des

Il faut maintenant nous opposer fermement à la réduction des dotations des CTI ! Sous réserve de l'adoption de ces deux importants amendements, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur les crédits de la mission « Économie

en matière de droit des entreprises et de droit de la consommation. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoyait initialement une diminution très forte des crédits de ce programme : 7,8 % de crédits de paiement en moins, pour un périmètre quasiment inchangé

En application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Autorité de la concurrence a rendu deux avis en matière de liberté d'installation des notaires. Dans le second avis, rendu le 31 juillet dernier, elle a proposé la nomination de 700 nouveaux notaires d'ici à 2020. Dans la mesure où 1 620 notaires viennent d'être nommés, au terme d'un lourd processus de tirage au sort, la question se pose de l'urgence, voire de l'utilité, pour le Gouvernement, de prendre un nouvel arrêté pour mettre en oeuvre cette dernière proposition.

Pour que cette administration assure pleinement sa mission de contrôle et de protection des consommateurs, il importe de recentrer ses activités et de réorganiser ses services déconcentrés. Madame la secrétaire d'État, ce chantier reste, à ce jour, largement ouvert. Je vous invite à être ambitieuse en la

essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur les services déconcentrés. Une telle évolution tire les conséquences du manque de moyens de l'État et de la montée en puissance des régions dans le domaine du développement économique local. Nous souscrivons à une telle démarche : il faut rationaliser le travail des acteurs chargés du soutien aux entreprises et du développement Madame la secrétaire d'État, ne peut-on aller plus loin dans la restructuration des services déconcentrés, pour améliorer davantage encore la cohérence des politiques d'accompagnement des entreprises dans les territoires, sous l'égide des régions ?

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je pourrais vous faire cinq minutes sur le désengagement de l'État sur cette mission, qui a vocation à soutenir les PME et l'industrie. Mais je préfère laisser la parole aux centaines de personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Comme Laurie, elles rêvent, madame la secrétaire d'État, de pouvoir vous raconter leur vie en direct. Je ne veux pas être leur porte-parole, je n'ai pas cette prétention. Je serai simplement leur voix ici, en lisant leur message. Et ils ont beaucoup à vous dire de leur souffrance, de leur colère, de leurs espoirs, qu'ils portent des gilets jaunes ou pas, qu'ils luttent ou qu'ils ne le puissent pas, en raison de leurs petits salaires ou de leur isolement. Par exemple, Amadou a un avis sur la mission que nous examinons aujourd'hui Ils ont donné 5 milliards aux riches en supprimant l'ISF, ils ont dilapidé 100 milliards d'euros de CICE, ils ont même accordé des exonérations fiscales aux londoniens, et ils laissent 80 milliards d'euros échapper au fisc Et ils disent qu'ils soutiennent les PME, les artisans et les petits ? » JM, lui, veut nous parler de la valeur travail : « Je suis un papa seul avec mon fils de treize je suis boucher de métier et je bosse 45 heures par semaine pour 1 998 euros par mois. Vous voyez, ce mois-ci, on est le 15 et je suis déjà à découvert. On va finir le mois en mangeant des produits du magasin où je bosse et dont la date de consommation est dépassée. Alors, je ne me plains pas, mais, voilà, c'est une réalité, le travail ne paie plus. » Claire ajoute, sur le commerce et l'artisanat : « Trouvez-vous normal que moi, qui ai un petit magasin de vêtements, je sois moins aidée proportionnellement que l'hypermarché à 30 Je travaille 50 heures par semaine, j'élève seule mon enfant et je ne m'en sors pas. Il ne reste plus que deux magasins dans ma petite ville des Landes. Si je ferme, c'est du lien social qui se perdra et une ville qui se mourra. » Madame la secrétaire d'État, il faudra expliquer à Claire pourquoi le Fonds d'intervention pour Pour parler d'industrie et d'emploi, je cède volontiers la parole à Fabrice : « Je suis chez PagesJaunes Solocal depuis dix-neuf ans. Depuis quelques années, je vois les profits de l'entreprise s'envoler, et les dirigeants se servir l'un après l'autre sur l'exécution sociale des salariés. Jour après jour depuis l'année passée, je vois les salariés partir en arrêt maladie, faire des tentatives de suicide, mourir à petit feu, comme mon entreprise, ce fleuron du digital français. Et je la vois abandonnée par l'État. Je la vois sombrer lentement vers les mains rapaces d'entreprises étrangères qui s'apprêtent à tuer le savoir-faire et les vies françaises qui y sont liées. Et je vois mon pays qui ne fait rien, qui nous laisse mourir, au nom du sacro-saint profit de quelques dirigeants ! Je vois la mort et l'État n'est pas là. C'est ça, la ? Pour servir seulement quelques dirigeants ? Le profit individuel au détriment de l'économie d'un pays est comme la pollution environnementale : c'est une intoxication. » Boris veut vous parler lui aussi de son entreprise, Alstom : « Je bosse comme ingénieur chez Alstom depuis décembre 2005. Nous concevons et fabriquons les trains et les équipements ferroviaires pour la mobilité efficace, sûre et peu polluante, tant pour les personnes que les marchandises. Et ce gouvernement laisse nos patrons donner l'entreprise au groupe Siemens, avec uniquement l'objectif de sortir du pognon Cette opération entraînera la braderie de nombreux sites, puis, comme ils disent, des " rationalisations ", avec suppressions de capacités et d'effectifs. Quand l'État français fera-t-il arrêter cette opération et développera-t-il une vraie stratégie industrielle pérenne pour la filière ferroviaire ? Enfin, pour conclure, je souhaite vous lire un mot de Sandra, qui nous interpelle toutes et tous : « Sachez que, du haut de mes vingt-quatre ans, j'ai peur pour mon avenir Que vais-je devenir ? Mes futurs enfants vont-ils encore pouvoir vivre ? Je me permets de vous écrire aujourd'hui, après ma longue journée de travail, pour vous poser une question toute simple : que puis-je faire à ma petite échelle pour essayer de changer tout ce qui se passe en ce moment ? indignez-vous ! Engagez-vous ! Nous avons besoin de toutes et tous pour bousculer l'ordre établi, faire en sorte que cette économie soit au service de l'humain et de notre planète, et non l'inverse.

en comparaison avec les budgets, par exemple, de l'éducation ou de la défense, et son périmètre change peu par rapport à 2018. Avec le léger ralentissement de la croissance économique constaté cette année et de fortes incertitudes pesant en particulier sur le commerce international l'an prochain, on voit le bien-fondé d'une telle politique publique et, en même temps, l'ampleur des défis auxquels elle doit répondre. La réduction des crédits l'an prochain correspond notamment à une rationalisation des dépenses d'intervention, environ 18 % des crédits de la mission, avec la diminution des aides aux PME du commerce et de l'artisanat. Pour ma part, je soutiens l'idée des rapporteurs spéciaux selon laquelle le transfert de compétences aux collectivités, en particulier aux régions, qui est tout à fait légitime,

mon groupe s'associe à la proposition des rapporteurs spéciaux de rétablir ses crédits à 30 millions d'euros. Nous allons même un peu plus loin dans la volonté de refinancement, en proposant d'augmenter ces crédits à 36 millions d'euros, en cohérence, en particulier, avec notre proposition de loi, adoptée par le Sénat le 21 novembre dernier, visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux. Je ne souhaite toutefois pas céder à un certain misérabilisme et j'en profite pour saluer des programmes tels qu'« Action coeur de ville », qui me paraît une excellente initiative gouvernementale En matière de politique commerciale, nos entreprises ont toujours un besoin criant de soutien à l'export. Nous devons beaucoup plus nous inspirer de l'exemple de nos voisins allemand et italien, qui comptent de nombreuses entreprises exportatrices, avec une balance commerciale nettement plus positive que la nôtre. La mise en place de « Team France Export », visant à mieux coordonner les actions de Business France, des chambres consulaires et des régions, est un pas dans la bonne direction. Encore faudra-t-il renforcer notre tissu industriel, structurellement

un délai de restriction budgétaire plus long, afin que les CCI puissent mieux préparer leur mutation. J'en viens maintenant au très haut débit. La couverture du territoire en très haut débit, dans le cadre du programme 343, reste un point d'attention. En la matière, un véritable enjeu d'aménagement du territoire, qui doit être plus étroitement associé à d'autres dimensions, comme la politique des transports, qui sera abordée prochainement, au travers du projet de loi d'orientation des mobilités, ou encore la politique du logement. Avec la première superficie d'Europe de l'Ouest, la France est un grand pays- pas seulement par la surface, d'ailleurs -, avec une population fortement concentrée en Île-de-France et dans les autres grands centres urbains, raison pour laquelle les questions d'aménagement, notamment d'aménagement du territoire, y sont plus aiguës qu'ailleurs. Enfin, en ce qui concerne la reprise d'entreprises, il paraît important de donner au Fonds de développement économique et social, le FDES, des marges de manoeuvre plus importantes, sans nécessairement recourir à la loi de finances. En effet, la rapidité des décisions est déterminante dans ce domaine. Les avances attribuées par l'État à des entreprises comme Presstalis ou Ascoval, même si elles ne représentent qu'une part limitée du financement de la reprise, peuvent constituer le « coup de pouce » nécessaire au succès de l'opération. C'est pourquoi le FDES doit avoir les moyens de se montrer le plus réactif possible. À cet égard, je ne suis pas favorable à ce que

la mission « Économie » rassemble les programmes et les administrations qui ont pour objet d'encourager l'emploi, la compétitivité, les exportations, la concurrence et la protection des consommateurs. Elle est composée de quatre programmes, dont le récent programme « Plan France Très haut débit qui devrait financer la couverture intégrale du territoire en internet fixe à très haut débit d'ici à 2022. Cette mission est stratégique à plus d'un titre. D'abord, elle doit être accompagnée d'une vraie réflexion sur le rôle de l'État dans l'économie. Un État stratège, dans une économie mondialisée, doit savoir associer volontarisme politique et libération des énergies. Il doit accompagner les mutations du monde du travail, sans laisser un seul travailleur au bord du chemin. du chemin. Nous ne pouvons pas nous résigner à la chute vertigineuse de l'emploi industriel que nous connaissons depuis quelques années. À cet égard, cette mission devrait être une mission de reconquête je crois profondément que, sans tissu industriel robuste, il n'est pas de puissance commerciale. Par exemple, les excédents titanesques de l'Allemagne sont le fruit de politiques de long terme pour renforcer le, le puissant réseau de petites et moyennes Si la France est encore le sixième exportateur mondial de biens et de services, pour un moment équivalent à près de 30 % de son produit intérieur brut, les chiffres du commerce extérieur ne sont pas à la hauteur des attentes depuis quelques années. Le solde des échanges de biens a baissé de près de 30 % en quatre ans. Le déficit commercial de la France s'est creusé continûment depuis le début de l'année et atteint 48 milliards d'euros sur neuf mois.

Je rappelle que la France ne compte que 125 000 entreprises exportatrices, la plupart étant de grands groupes et des ETI. En Allemagne, ce chiffre atteint 350 000, avec une majorité de PME. Nous devons prendre en compte ce retard criant, dont le comblement devrait être une priorité. Ce sont les grosses PME et les ETI qui peuvent nous faire gagner des parts de marché à l'international.

Nous rejoignons le Gouvernement quant à sa volonté de mettre le patrimoine de l'État au service de la reconquête industrielle et de l'innovation, mais nous serons vigilants sur le suivi des cessions d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux. Nous ne voulons pas d'un bradage des intérêts patrimoniaux de l'État. Il faudra que les sommes levées abondent réellement le fonds pour l'innovation et l'industrie et que celui-ci soit utilisé à bon escient. Pour terminer, je m'attarderai sur le plan France Très haut débit. Lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, le Président de la République s'est engagé sur l'objectif d'une couverture du territoire en haut débit d'ici à 2020 et en très haut débit d'ici à 2022. Aujourd'hui, soit un an et demi plus tard, il semble que nous sommes assez loin du compte pour la France rurale : seuls 31,2 % des ménages et locaux professionnels ont accès au très haut débit La réussite du plan est pourtant essentielle pour nos concitoyens, pour nos entreprises et pour l'accès à des services publics de plus en plus dématérialisés. Pour conclure, l'effort sur les crédits de cette mission stratégique pourrait être plus important. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut mieux évaluer les aides aux entreprises et ne pas les saupoudrer, mais les crédits attestent d'un manque d'ambition pour nos PME. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, 82 %, c'est la proportion d'entreprises étrangères qui jugent que la France est un pays où il faut investir en 2018, contre 23 % en 2014. Non seulement l'opinion des investisseurs étrangers sur la France s'améliore, mais, en plus, leurs intentions se concrétisent. Il faut le dire, les chiffres de l'attractivité et des investissements étrangers en France sont les meilleurs depuis deux quinquennats : le nombre d'investissements industriels étrangers en France a bondi de 52 %. Pourtant, il reste beaucoup à faire pour renforcer la compétitivité de notre pays. je dis « compétitivité », il ne faudrait pas que les plus interventionnistes d'entre nous entendent « thatchérisme » ou pensent au scénario d'un film de Ken Loach. « Compétitivité » ne signifie pas dérégulation, abandon du politique au profit de l'économie, services publics vendus. J'en veux pour preuve que les classements mondiaux placent la France après la Finlande ou la Suède, pays dont on ne peut pas dire qu'ils aient des services publics déficients. Les mesures qui constituent la stratégie économique du Gouvernement dessinent un modèle plus durable, plus efficace, plus attractif- en fait, plus en phase avec l'économie du XXI siècle. Il s'agit tout d'abord de transformer notre modèle fiscal, en diminuant la fiscalité du capital et celle qui pèse sur les entreprises. Ce sujet a été abandonné par la majorité sénatoriale, qui n'en parle jamais, mais les prélèvements obligatoires sur les entreprises baissent, cette année, de 19 milliards Le crédit d'impôt recherche est sanctuarisé, des suramortissements sont mis en place pour les dépenses d'innovation, la fiscalité du capital est allégée. Ces décisions s'expliquent par une raison simple : nous sommes dans l'économie du numérique, et celle-ci a besoin de capital. Or on compte 133 robots en moyenne par habitant en France, contre 190 en Italie et plus de 300 en Allemagne pour renforcer la compétitivité des entreprises, il faut aussi des efforts de rationalisation, car il n'y aura pas de croissance durable sans réduction des dépenses publiques. C'est le sens de la trajectoire de baisse de la fiscalité affectée aux chambres de commerce et d'industrie.

plutôt qu'aux coups de rabot antérieurs. En parallèle, on baisse la fiscalité sur les entreprises. Cela est cohérent. Mieux faire, c'est aussi réformer la présence de l'État. Le programme 134 présente une refonte de la présence territoriale et des missions des conseils, directions et autorités administratives indépendantes, à l'image de la présence de la direction générale des entreprises en région, dont la mission est clarifiée : elle se voit chargée de l'accompagnement des entreprises en difficulté, du développement des filières stratégiques et du soutien à l'innovation. marque aussi un tournant. Il est temps de prendre des décisions claires et de les expliquer. Les décisions sont acceptées si elles sont justes ! Les Français ne veulent pas moins de services publics lorsqu'ils demandent moins d'impôts

si le chômage a persisté à des niveaux élevés, c'est qu'il n'y avait pas de majorité politique pour une réforme du marché du travail. Que fait le Gouvernement ? Il agit sur le marché du travail.

! Réduire les trappes à chômage et à pauvreté, c'est aussi valoriser le travail. Avec l'augmentation de la prime d'activité, c'est un budget de 6 milliards d'euros qui est sanctuarisé. Enfin, la compétitivité ne signifie pas des services publics au rabais. Elle implique, au contraire, des « services publics du XXI siècle » ! Les décors de la salle des conférences du Palais du Luxembourg, où siège le Sénat, nous rappellent les progrès du XIX siècle, notamment l'électrification du territoire.

est territoriale. Le programme 343 de la mission « Économie » porte la couverture du territoire en très haut débit à 100 % d'ici à 2022. Ce plan est couplé à une accélération du déploiement de la 4G. Malgré les critiques sur les plans successifs, le manque de moyens ou la stratégie menée, qui ne correspondait pas aux réalités des territoires,

Mes chers collègues, si l'avenir est imprévisible, il se prépare. Il se prépare avec une stratégie claire, cohérente, tournée vers la création de valeurs et vers l'emploi. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais utiliser les quatre petites minutes qui m'ont été allouées pour aborder la question importante de la stratégie industrielle de l'État, qui devrait être au coeur des crédits de la mission « Économie », et je vais le faire en évoquant une opération à 10 milliards d'euros. Dans leur récent rapport d'information, nos collègues Martial Bourquin et Alain Chatillon appellent l'État à renouveler sa vision stratégique en faveur de l'industrie. Nous souhaitons, avec eux, la redynamisation de l'outil actionnarial de l'État. Dans ce cadre, la vente d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des jeux nous paraît un mauvais choix,

cette opération est opaque et aucune explication fournie jusqu'ici par les membres du Gouvernement interrogés n'a été de nature à nous convaincre de sa pertinence. Contrairement à ce qui a été annoncé au départ, ce ne sont pas 10 milliards d'euros qui vont être affectés au soutien à l'innovation, mais le produit des dividendes générés par le placement des actions que vous allez vendre.

Certes, vous allez réintégrer immédiatement 10 milliards d'euros, ce qui vous évitera peut-être de passer le cap symbolique des 100 % de PIB de dette publique. Mais quelle est la vraie logique de cette opération de vente et d'abandon de fleurons nationaux ? À qui profite-t-elle vraiment ? Dans ces conditions d'incertitude et de risques, nous ne sommes pas favorables à ces privatisations. Pour éviter de revivre la calamiteuse opération de 2005 concernant les autoroutes, il faut que le produit des ventes de ces trois entreprises soit au moins égal à la somme, actualisée sur la très longue période, du produit des dividendes auxquels l'État va renoncer. À cet égard, comment comptez-vous procéder et quels sont vos objectifs ? Rien dans les crédits de la mission ne nous permet de l'appréhender. Toujours sur ce sujet des privatisations, vous avez annoncé envisager de monter au capital d'EDF dans le cadre de la donne nouvelle qu'induit la programmation pluriannuelle de l'énergie et la montée en charge indispensable des énergies renouvelables. La grande entreprise qu'est EDF ne doit pas être sacrifiée comme l'ont été d'autres secteurs de la production industrielle française dans le passé. Ce qui s'est passé avec Alstom et AREVA, par exemple, nous fait craindre l'amorce d'un démantèlement de la filière nucléaire intégrée française. Il y va de notre souveraineté nationale, du rôle et de la place géopolitique de la France en Europe et dans le monde de l'énergie. Il y va aussi du savoir-faire de très haut niveau des titulaires de centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Faute, à ce stade, de clarté dans votre stratégie, les inquiétudes sont fortes. Va-t-on vers un démantèlement de l'entreprise, aujourd'hui intégrée, et une revente à la découpe ? Je pense, par exemple, à RTE. Quelle place reviendra aux énergies renouvelables, à côté du nucléaire et de l'hydraulique ? Et, en lien direct avec le budget pour 2019, quel sera le niveau des nouvelles prises de participation et comment seront-elles financées dans le contexte que nous constatons, celui d'un endettement fort qui continue à s'accroître tendanciellement ?

comme la plupart des pays développés, la France a été confrontée, ces dernières décennies, à la désindustrialisation de son économie, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut passant de 24 % en 1980 à 12,6 % en 2016. Depuis l'an 2000, 25 % de l'emploi industriel a disparu. Si ce Si ce phénomène a plusieurs origines, l'État doit se donner les moyens d'accompagner efficacement son industrie et les territoires et se comporter en véritable stratège. ce projet de loi de finances a de quoi nous laisser dubitatifs. Sous couvert de rationalisation des aides aux entreprises, la tendance constatée par l'ensemble de nos rapporteurs est celle d'un désengagement de l'État. En effet, si les engagements du plan France Très haut débit sont à saluer, ils doivent néanmoins être accélérés, et de nombreuses inquiétudes perdurent par ailleurs. Les autorisations d'engagement chutent de 17 % par rapport à 2018. Près de la moitié des crédits de la mission sont désormais consacrés à des dépenses de personnel. Moins d'un euro sur trois est réellement dédié à des dépenses d'intervention.

Que comprendre de la gestion extinctive du FISAC, alors même que celui-ci constitue un outil d'intervention ponctuelle et ciblée, dans un objectif de rééquilibrage et de complémentarité avec les actions locales ? nous saluons bien évidemment la position de la commission des affaires économiques et soutiendrons l'amendement tendant à abonder les crédits du FISAC de 30 millions d'euros en autorisations d'engagement. Derrière ces éléments, il y a bien la crainte que l'État stratège ne soit pas au rendez-vous. Or notre stratégie industrielle en dépend. Nous devons marcher sur nos deux jambes, à savoir l'investissement et le fonctionnement,

je vous proposerai d'adopter un amendement visant à abonder ce fonds, qui est un outil complet, permettant, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de favoriser le développement économique et social d'une aire géographique et de soutenir des projets modernes, innovants et préparant la restructuration industrielle de la filière de l'acier. Ascoval en est

d'État, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par les rapporteurs sur la mission « Économie » du projet de loi de finances pour 2019. J'entrerai rapidement dans le vif du sujet : comment examiner ce projet de budget sans le relier à l'actualité, sans faire le lien avec ce qui se passe dans nos départements ?

Élue d'un territoire rural et de montagne, les Hautes-Alpes, comment pourrais-je ne pas revenir sur le désengagement de l'État dans les actions territoriales qu'il devrait conduire en faveur des entreprises et des consommateurs ? C'est aussi pour cette raison que nos concitoyens manifestent : parce que la spécificité des territoires n'est pas prise en compte et que, notamment, en zone rurale, aucune réponse n'est apportée, aucune solution n'est trouvée. Prenons l'exemple du FISAC. Ce dispositif a été créé en 1985 pour soutenir les services de proximité, menacés ou fragilisés par la désertification dans les espaces ruraux et pour remédier aussi à la dévitalisation des centres-villes. En 2019, seuls 6,1 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus au bénéfice d'opérations ayant fait l'objet de décisions de subventions au cours des années précédentes. Malgré la réforme de 2014 censée relancer le dispositif, les montants engagés n'ont cessé de diminuer, de 80 % entre 2010 et 2018. territoriale de la République, doit nous conduire à nous interroger sur certains dispositifs eu égard aux compétences désormais dévolues aux collectivités territoriales, l'État ne doit pas, pour autant, se désengager des actions économiques de proximité. En effet, je crois, au contraire, que l'État doit s'assurer d'un rééquilibrage économique territorial. C'est pourquoi il doit maintenir des interventions ciblées. C'est d'ailleurs l'objet principal du FISAC, qui a non pas vocation à se substituer aux régions, mais plutôt à agir en complément, voire en dernier recours. Ce dispositif porté par l'État est d'autant plus nécessaire que de nombreuses communes rurales voient leurs dotations baisser du fait de la recomposition de la carte intercommunale, ce qui limite considérablement leur capacité d'intervention. Si l'on peut se réjouir de la mise en oeuvre du plan « Action coeur de ville », il ne peut être l'unique réponse à l'ensemble des problèmes de dévitalisation, puisqu'il ne vise pas les mêmes opérations que le FISAC

La suppression du FISAC vient également remettre en cause les engagements pris par le Gouvernement en faveur des stations-service de proximité, sans qu'il soit proposé de solution alternative. Au travers de l'actualité, on mesure à quel point il s'agit pourtant d'un enjeu crucial pour la cohésion de nos territoires ruraux. Enfin, je voudrais revenir aussi sur la compétitivité des entreprises et l'ambition annoncée par le Gouvernement de favoriser un environnement économique propice à la croissance et à l'emploi. En effet, les risques de voir disparaître les chambres de commerce et d'industrie hyper-rurales sont importants, puisque la réduction de la taxe affectée au réseau CCI France est une réalité. S'il appartient aux CCI de région de procéder annuellement à la répartition de la taxe pour frais de chambre et d'ajuster le montant attribué à chacune des CCI, la situation de celles qui sont situées en zone hyper-rurale doit faire l'objet d'une attention particulière. Leur rôle est essentiel pour le tissu économique local, car elles assurent un accompagnement de qualité que les petites entreprises, voire les très petites entreprises, ne pourraient se payer. Dans ce contexte et au regard de leurs spécificités, de leurs besoins et de leur dépendance à la ressource fiscale, il me paraît indispensable qu'un régime dérogatoire puisse être étudié au bénéfice des CCIT, les chambres de commerce et d'industrie Vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations demeurent à ce stade. J'espère que nos discussions seront de nature à répondre aux attentes des entreprises, notamment dans les territoires ruraux. La parole

une loi destinée à sauver nos centres-bourgs et nos centres-villes d'un péril, d'un désastre. Le Sénat, cette assemblée des territoires, était légitime à le faire. Voyez en notre voix celle de ceux qui n'en ont pas, hélas ! Voyez en notre voix celle des maires de villes, de toutes les villes, car aucune n'est épargnée ! Voyez aussi en notre voix celle des milliers de commerçants ! Il est temps d'agir. De quoi s'agit-il en fait ? Ce que l'on peut considérer comme un outil de progrès, internet,- et je partage cet avis -programme une cyberéconomie, qui est devenue un péril pour le commerce des villes. Ne voyez surtout pas en moi une ringarde qui vivrait sur une autre planète Des magasins sont condamnés à fermer ; des rues entières sont réduites à un. Pis, le vivre-ensemble, ces rencontres souvent heureuses entre générations, au hasard d'un parc, d'un jardin public, d'une boutique, se meurt. Dans le confort du canapé, avec la facilité d'un clic, de la touche « Validez votre commande », le commerce se fait ailleurs : ailleurs, autrement, on ne sait même pas où En attendant chez nos compatriotes une véritable prise de conscience autour d'un acte d'achat conscient, doit-on accepter la facilité du pot de terre contre le pot de fer ? Doit-on accepter sans sourciller que ce qu'il est convenu d'appeler les GAFA- Google, Amazon, Facebook Apple -, auxquels on rajoute maintenant un « M » pour Microsoft, tuent à petit feu tous les jours ce qui fait notre humanité ? Ces grands groupes, à la santé insolente et aux profits qui grimpent à une vitesse vertigineuse, doivent contribuer au maintien tout simplement de la vie- oui, de la vie ! -et au maintien de l'emploi dans les villes, à tous ces métiers : il faut redonner de la lumière bienfaisante à nos vitrines, de la chalandise et de l'activité. Ces grands groupes, au moyen de toute espèce d'astuces fiscales, y compris d'odieux chantages aux États, se doivent de contribuer au retour de la vie. Il est urgent d'agir. Il sera courageux d'agir. Vous le savez, le courage est d'ailleurs cette belle valeur, cette inestimable valeur qui doit sous-tendre toute action politique. La

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, ce projet de loi suit le cap fixé par le Gouvernement : construire une prospérité qui doit bénéficier à tous les Français et à tous les territoires, une prospérité qui doit reposer non pas sur plus de dépense publique et, par conséquent, plus d'impôts, mais sur plus d'activité et, par conséquent, plus d'emplois pour les Français et pour leur entreprise. Je dois dire que cet objectif me semble d'une brûlante actualité. Je suis d'accord pour dire qu'il faut aussi du courage pour mener cette baisse des dépenses publiques et essayer de soutenir nos entreprises,

industrielle- on parlera de politique industrielle -et à l'export. Si les résultats sont là depuis mai 2017, ils ne sont pas suffisants, nous en sommes d'accord. Nous devons accélérer la transformation économique que nous menons. Certes, plus de 200 000 emplois ont été créés en un an.

L'économie française a notamment du retard dans deux domaines, comme vous l'avez souligné, la robotisation et la numérisation, et elle n'est pas en pole position en matière d'innovation de rupture.

Elle sera complétée à partir de 2020 par une baisse des taux. Là encore, cette mesure bénéficiera aux entreprises. Cette réforme vise, d'une part, à mettre en place un nouveau modèle pour les CCI afin que celles-ci se concentrent sur leur coeur de mission : assurer l'appui aux entreprises, la formation initiale et la représentation des entreprises. Elle tend, d'autre part, à alléger les impôts pesant sur la compétitivité des entreprises. Dans ce cadre, des mesures d'accompagnement importantes sont d'ores et déjà prévues par la loi PACTE : on ne laisse pas les chambres de commerce et d'industrie sans rien. Trop sympa ! D'autres mesures contribuent à la baisse de la pression fiscale dans le projet de loi de finances pour 2019. Ainsi, le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, est transformé en allégement de charges pérennes,

essentiellement du basculement d'un financement par crédit budgétaire à un financement par taxe affectée pour le CTI de la fonderie. Il ne faut donc pas surinterpréter les chiffres. En matière industrielle, nous souhaitons également nous attaquer aux impôts de production, qui minent la compétitivité de nos entreprises. D'importantes décisions ont déjà été prises par le Gouvernement, lesquelles conduiront à des des baisses d'impôt sur la production ; cette mesure concerne clairement les entreprises industrielles. Au total, l'ensemble de ces mesures réduira les impôts de production de plus de 1,5 milliard d'euros d'ici à la fin du quinquennat. C'est une première réponse à votre préoccupation en matière industrielle, monsieur Bourquin. Au-delà des mesures qui ont déjà été décidées, sachez que nous continuons à explorer le sujet, car il faut effectivement aller plus loin. Cela ne suffit évidemment pas. Nous devons en parallèle, par comparaison avec nos voisins européens, améliorer notre compétitivité hors coûts. Pour ce faire, nous devons impérativement miser sur l'amélioration de notre appareil productif. C'est pourquoi nous investissons massivement dans l'innovation. Nous avons sanctuarisé le crédit d'impôt recherche. Nous avons également augmenté les crédits en faveur du dispositif « Jeune entreprise innovante », dont l'efficacité économique a été largement démontrée. Par ailleurs,

On garantit ici la capacité d'investir 250 millions d'euros dans des innovations de rupture, l'intelligence artificielle et le stockage des énergies renouvelables, par exemple. Investir, c'est également numériser et robotiser les PME industrielles. Le dispositif de suramortissement que nous mettons en place répond à cet enjeu. Concrètement, cela représentera une baisse pouvant aller jusqu'à 11 % du coût de l'investissement, par exemple dans des imprimantes 3D, des capteurs connectés ou encore des robots. De manière plus générale, je veux faire observer que la politique industrielle ne se résume pas à la mission « Économie » ni au service de la DGE. En témoigne le dispositif « Territoires d'industrie », qui mobilise plus de 1,3 milliard d'euros de crédits dédiés.

sur lesquels on pourra revenir. Enfin, pour la première fois, la mission « Économie » alloue 175 millions d'euros de crédits de paiement au programme « Plan France Très haut débit », manifestant notre engagement sur ce sujet.

L'action publique doit aussi être plus efficiente et plus proche du terrain ; je ne pense pas que vous me contredirez ... Le ministère de l'économie et des finances se doit évidemment d'être exemplaire sur ce point. Nous avons donc décidé de transférer ou de fusionner les dispositifs qui ne relèvent plus de l'État et qui ne sont plus portés aujourd'hui par des acteurs les mieux placés pour être efficaces. Le FISAC, auquel le Sénat est, je le sais, très attaché, ne financera plus de nouveaux projets. Cette décision nous semble cohérente avec la compétence donnée aux régions en matière de développement économique depuis la loi NOTRe. Elle s'inscrit dans l'application de la loi et va dans le sens d'un renforcement des compétences des régions et des collectivités, qu'un certain nombre d'entre vous appellent de leurs voeux. Cela ne signifie pas la fin d'un accompagnement ; ce sera la mission de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Dans cette même logique d'efficacité et de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, nous allons engager, vous l'avez souligné, une réforme ambitieuse de la direction générale des entreprises, qui sera recentrée sur ses missions stratégiques : accompagnement des entreprises en difficulté, desquelles les PME industrielles ; développement des filières stratégiques et de l'innovation, avec, notamment, la participation aux instances de gouvernance des écosystèmes d'innovation. Cette évolution impliquera de réduire les effectifs du réseau déconcentré de la DGE de 330 ETP, ou équivalents temps plein, une baisse qui s'étalera sur trois ans, avec un accompagnement particulier. Nous avons par ailleurs entamé, comme vous l'avez souligné, monsieur Lalande, une réforme du dispositif de soutien à l'export : elle vise à rationaliser l'action des divers acteurs publics concernés afin de renforcer la lisibilité et l'efficacité du dispositif d'accompagnement. En France, un guichet unique « Team France Export » sera mis en place dans chaque région, réunissant Business France et les chambres de commerce et d'industrie, dont la mission est d'identifier et de préparer les entreprises à l'export. En parallèle, les correspondants uniques de « Team France Export » seront mis en place à l'étranger. Cette réforme s'achèvera au début de 2019.

Cette stabilité des crédits traduit notre volonté de mieux cibler les aides et de les rendre plus efficaces, afin d'améliorer l'efficience de notre gestion publique. La parole

les vôtres ! -montrent que la dépense publique, en particulier la dépense de l'État, continue d'augmenter ! Très peu ! Ne commencez pas votre propos par des provocations à l'encontre du Sénat. Nous sommes plutôt dans

Entre 2010 et 2018, la dotation du FISAC est passée de 64 millions d'euros à 16 millions d'euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans,

Malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l'année dernière pour préserver cet outil précieux afin de lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer. Ce désengagement de l'État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient, par ailleurs, leurs dotations diminuer du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale. Surtout, cet amendement s'inscrit dans la démarche du groupe du RDSE pour donner les financements nécessaires au dispositif de la proposition de loi, portée par Éric Gold, adoptée par le Sénat le 21 novembre 2018, visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux.

pour lui permettre d'atteindre 30 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisation d'engagements, alors que le projet de loi prévoit seulement des crédits de paiement à hauteur de 6,1 millions d'euros et aucune autorisation d'engagement. Sur ces 30 millions, 5 millions d'euros seraient réservés au financement des stations-service indépendantes. En effet, le maintien du FISAC, doté d'un montant suffisant, est indispensable à l'heure où le Gouvernement entend faire de la redynamisation commerciale une priorité. La situation des stations-service de proximité doit, quant à elle, faire l'objet d'une attention particulière.

Cet amendement vise à rétablir les crédits du FISAC à hauteur de 30 millions d'euros.

pour atteindre 30 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement, alors que le projet de loi prévoit seulement des crédits de paiement à hauteur de 6,1 millions d'euros et aucune autorisation d'engagement. Entre 2010 et 2018, la dotation de ce fonds est passée de 64 millions d'euros à 16 millions d'euros, soit une baisse de 80 %. Pourtant, nous sommes nombreux ici et sur toutes les travées à nous accorder à dire que le FISAC est l'un des outils, de moins en moins nombreux, dont disposent encore les élus locaux pour redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. Cela étant, cette redynamisation doit être globale et exige que l'on mette en place, dans le même temps, d'autres actions, en particulier en ce qui concerne l'habitat et l'accueil de nouvelles populations. Le FISAC existe et il ne doit pas être un simple outil d'accompagnement de l'austérité dans nos territoires ruraux. Au contraire, il joue un rôle essentiel pour préserver et développer le tissu des entreprises de proximité, qu'elles agissent dans le domaine du commerce, des services ou de l'artisanat. Il participe également pleinement à l'objectif fondamental de lutte contre la désertification commerciale des zones rurales, à laquelle nous sommes ici toutes et tous attachés et il doit être- j'ai même envie de dire : il doit rester -l'un des leviers permettant de faire République, un des leviers permettant de garantir l'égalité républicaine pour tous nos

d'une volonté de se désengager, il s'agit tout simplement de la volonté d'éviter les doublons et de fonctionner main dans la main avec les régions -des nouvelles missions économiques des régions.

y compris dans les petites communes. C'était un soutien très important. Évidemment, 30 millions, ce n'est pas 200 millions, ni 600 millions, ni des milliards, comme on les manie ici dans le budget, mais, pour les maires des petites communes, ce sont des soutiens extrêmement efficaces à des actions extrêmement modestes, mais qui sont structurantes pour notre tissu rural.

mais quelle expérience avez-vous des territoires ? Quelle expérience avez-vous de ce que vit un maire lorsqu'il cherche tout simplement à sauver l'économie de son village ? On nous a déjà supprimé la réserve parlementaire.

les maires passent leurs journées à contractualiser sans que l'État apporte ensuite les contributions nécessaires. Il est vraiment extrêmement important de revoir la façon dont vous envisagez les aides aux territoires.

qui participent à l'équipement des territoires. Or on sait que la plupart des projets financés par le FISAC ou d'autres dispositifs sont réalisés concrètement par des artisans.

entre la première partie et la deuxième partie de la loi de finances, entre la dépense publique, en général, et les dépenses publiques, en particulier. Je ne sais

vous nous dites que le FISAC est inadapté, allez jusqu'au bout : inadapté à quoi ? Inadapté à la ruralité ? Inadapté aux communes rurales ? Inadapté aux services de proximité ? Allez jusqu'au bout, dites carrément qu'il faut supprimer les communes et ne pas s'occuper de la ruralité

vous disent tous la même chose, que vous pourrez longtemps avoir raison toute seule, au nom d'une expertise sur laquelle vous n'êtes même pas capable de vous exprimer ? Quand M. Bargeton nous

banlieues, est malvenu ! Ceux qui sont déconnectés aujourd'hui, ce sont ceux qui sont aux manettes, et les Français vous le disent tous les jours

c'est la rue, le village, c'est le centre-bourg, c'est l'ancien chef-lieu de canton- bien qu'on ne sache plus très bien ce que sont les chefs-lieux de canton, mais ça existait et c'était extrêmement important. Alors, c'est certain

-, d'une évolution qui pèse aujourd'hui sur notre capacité à retrouver une trajectoire des finances publiques qui soit soutenable.

bien à cela que doit servir l'Agence nationale de la cohésion des territoires ! Je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement n'a pas une préoccupation pour les territoires. Toute la démarche des territoires d'industrie, qui est complète, consiste

avant de proposer un amendement à l'Assemblée nationale visant à « rétablir une ligne symbolique de crédits au sein du programme 134 afin de maintenir un [ ...] cordon ombilical reliant cette institution financière à la représentation nationale nationale ». Ce rôle de Bpifrance mérite plus qu'un cordon ombilical ! Il est d'autant plus essentiel que, si la distribution du crédit bancaire aux PME est satisfaisante, le taux d'accès au crédit des TPE reste toujours plus difficile, faute de garanties suffisantes à présenter par ces dernières. Même si un contexte économique à nouveau plus porteur permet d'envisager que les banques acceptent de prêter à l'avenir, en réduisant quelque peu le niveau de leur garantie, l'existence d'un mécanisme de garantie de masse sur fonds publics relativement robuste reste essentielle pour porter une économie en croissance. Il importe donc que Bpifrance conserve de réelles capacités d'action, en particulier à l'égard des TPE et PME. Entre 2013 et 2016, grâce à son activité de garantie, la banque a effectivement contribué à la mise en place de 24,2 milliards d'euros de financement, soutenant près de 640 000 emplois. Compte tenu des contraintes de transferts de crédits, cet amendement tend donc à minorer l'action n° 02, Développement international de l'économie française, du programme 305 de 29,8 millions d'euros, pour ramener l'action n° 20 du programme 134 à hauteur des crédits effectivement consacrés en 2018 à cette activité, soit 39,8 millions d'euros.

Chaque année, l'État verse une subvention à Bpifrance au titre de ses activités de garantie. Si cette subvention est supprimée en 2019, c'est, non pas parce que l'État se désengage

». Il consacre ainsi l'objectif du Gouvernement, rappelé lors de l'installation du conseil interministériel du tourisme, le 26 juillet 2017, de conforter la France dans sa place de première destination touristique mondiale, en portant le nombre d'arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l'horizon de 2020.

secteur du tourisme ont été transférés, à partir de 2014, au ministère de l'Europe et des affaires étrangères et ne relèvent plus de la mission. Je vous propose donc, ma chère collègue, de retirer votre amendement. Ce débat pourra avoir lieu, lors de l'examen en séance de la mission « Action extérieure de l'État

avis. Cet amendement de la commission des affaires économiques tend à maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire consacrée au soutien à la compétitivité des entreprises industrielles.

particulièrement, les PME pour 3,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et 4,98 millions d'euros en crédits de paiement. Le choix de privilégier des actions menées en partenariat avec les régions et les CCI est louable, mais il ne peut avoir pour effet de diminuer l'enveloppe globale des moyens consacrés à la compétitivité des entreprises industrielles. Par exemple, l'enjeu des pôles de compétitivité est essentiel. Le Gouvernement entend pourtant réduire fortement leur financement d'ici à 2022, ce qui conduirait à leur disparition. L'amendement de la commission vise donc à augmenter la dotation budgétaire consacrée aux actions pilotées de manière décentralisée, en y reportant le montant dédié, en 2018, aux actions pilotées en central. Ainsi, l'enveloppe globale des actions menées restera inchangée par rapport

Cette diminution de plus de 10 % des crédits, justifiée par un objectif global de maîtrise des dépenses publiques, remet en cause l'indépendance de ces associations. Nous proposons donc d'augmenter légèrement les crédits d'intervention pour la protection économique du consommateur, dans le but de les remettre au niveau de 2017. Pour ce faire, nous souhaitons majorer les crédits de l'action n° 24 du programme 134, « Développement des entreprises et régulations », de 1,4 million d'euros, somme qui serait transférée de l'action n° 01 du programme 305, « Stratégie économique et fiscale du programme 134 concerne les dépenses d'intervention à destination de l'Institut national de la consommation, l'INC, de quinze associations de consommateurs, du Centre européen des consommateurs France et du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. L'indépendance de ces organismes de protection des consommateurs vis-à-vis du monde économique est fondamentale. Elle leur permet d'informer, de conseiller et d'aider les consommateurs, dont elle représente les intérêts. Or, cette indépendance est garantie par les financements publics. C'est pour cette raison, mes chers collègues, que nous vous proposons cette majoration. L'amendement

à leur niveau de 2018. En effet, avant d'envisager une nouvelle réduction du montant des subventions disponibles pour l'écosystème de la consommation, il convient de procéder à un réexamen global de son organisation et du rôle respectif de chacun des intervenants. Dans l'attente des résultats de ce réexamen, auquel la commission des affaires économiques entend procéder prochainement, il est proposé, par cet amendement, non pas d'augmenter, comme dans l'amendement du groupe CRCE, mais de maintenir le montant des crédits aux acteurs de la consommation.

elle est aujourd'hui trop dispersée, entre quinze associations nationales et le Centre européen des consommateurs. Cela emporte deux conséquences majeures. Il y a redondance dans les activités conduites par ces acteurs, notamment en matière d'information du consommateur, puisque tous ont un site internet et la plupart des publications papier, et en termes de formation des personnels,

Ces différents éléments étaient à l'origine d'une utilisation des crédits publics, qui, insatisfaisante, ne pouvait pas perdurer, alors qu'il existe des gisements de synergies dans les territoires dont les subventions ont été préservées. Cette démarche a été comprise des associations de consommateurs les plus modestes, puisque trois d'entre elles préparent pour 2019 leur fusion et la création d'une nouvelle association les regroupant, ce qui leur permettra d'optimiser la mutualisation de leurs moyens et, surtout, d'améliorer leur présence sur le territoire.

méritent d'être soutenus. Notre amendement est simple : il vise à maintenir le niveau actuel de dotations budgétaires des centres techniques industriels et des organismes assimilés.

donnez-nous les éléments ! Nous n'avons rien à ce sujet. Nous devons maintenir la dotation budgétaire des CTI ; leur action est, selon nous, cruciale pour les PME industrielles. Ils diffusent, comme cela a été dit hier, le progrès technique et l'innovation auprès des entreprises de leur branche et les accompagnent dans la mise en oeuvre de leur modernisation. L'étranglement de leur financement serait lourd de conséquences pour le développement de nos entreprises, en particulier dans les territoires, y compris dans les territoires ruraux. Nous sommes donc convaincus qu'il est nécessaire- c'est l'objet de cet amendement -de conserver la dotation budgétaire des CTI à leur niveau de 2018, c'est-à-dire 9,95

Vous proposez donc de rétablir ce financement au même niveau que celui de l'an passé, à savoir 9,95 millions d'euros. Cependant, l'outil budgétaire n'est pas forcément le bon vecteur dans la mesure où le financement des CTI et des CPDE par subvention budgétaire a été progressivement remplacé par un financement au moyen de taxes affectées, suivant en cela la préconisation formulée en 2014 dans un rapport de Claudine Valter.

parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud. Le Président de la République a lancé un grand chantier de la transformation numérique de notre pays afin de rendre accessible le numérique à tous nos concitoyens et de couvrir l'ensemble de nos territoires. Nous disposons de plusieurs leviers pour porter cette pour porter cette politique publique. La Commission supérieure du numérique et des postes, ou CSNP, initiée par le président Larcher en 1990, fait partie de ces outils. outils. Parmi ses missions, la commission veille au bon déploiement de la couverture mobile et du très haut débit, ainsi qu'au développement de la cybersécurité. Elle exerce aussi un contrôle sur les opérateurs s'agissant de ses missions de service public. Composée de sept députés, de sept sénateurs et de trois personnalités qualifiées, la commission est placée auprès du Gouvernement. Elle est ainsi l'autorité politique du secteur du numérique et des postes. Ses moyens de fonctionnement, alloués par le ministère de l'économie et des finances, sont aujourd'hui éparpillés et peu lisibles. Aussi, afin de garantir la mise en oeuvre des interventions de la commission dans une période où le secteur du numérique est fortement sollicité, il serait souhaitable que son budget soit rassemblé dans un même programme. C'est l'objet de cet amendement. Il s'agit aussi de sanctuariser ses moyens à hauteur de 1 million d'euros, pour permettre à ses membres d'appréhender pleinement et en toute indépendance la place nouvelle du numérique dans les territoires et sur le plan international. Bonne idée ! Quel est l'avis de la commission ?

le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'échéance de 2022. Au total, l'investissement global se monte à plus de 20 milliards d'euros, dont la majeure partie est assumée par le secteur privé.

le cas échéant en lien avec un prestataire privé, l'État apporte à ces dernières son concours financier pour permettre d'atteindre l'équilibre financier des projets. Il s'agit d'assurer l'égalité d'accès au très haut débit en garantissant le raccordement au réseau, y compris dans les zones les moins denses. C'est une action d'aménagement du territoire. Afin d'aider les dernières collectivités à financer leur réseau, ou à le compléter, il est nécessaire que l'État puisse continuer à proposer des aides, un guichet dédié de l'Agence du numérique. Ce guichet a malheureusement été fermé en début d'année. L'Agence estime à environ 700 millions d'euros le besoin de financement résiduel nécessaire sur les années à venir afin de finaliser le réseau fibré. Par conséquent, il est proposé d'ouvrir dès cette année 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement, ce qui contribuera à adresser un signal aux collectivités et aux opérateurs et permettra d'engager de nouveaux projets. Le solde de l'investissement pourrait être prévu dans le projet de loi de finances pour 2020.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Dans le cadre de la refonte des droits et contributions perçus par l'Autorité des marchés financiers, le présent amendement vise, premièrement, à plafonner le taux de l'ensemble des contributions pour lesquelles le taux est fixé par décret, afin de garantir leur constitutionnalité ; ; deuxièmement, à exclure les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement de la contribution due en cas d'émission de parts sociales, dès lors que ces dernières sont déjà soumises à une contribution sur la base de leurs encours ; troisièmement, enfin, à apporter diverses corrections et précisions rédactionnelles.

duquel l'Autorité des marchés financiers est autorisée à percevoir des « contributions volontaires » versées

On pourrait d'ailleurs remplacer tous les impôts par des contributions volontaires, mais je ne suis pas sûr que cela marcherait ... L'objectif sous-jacent consistait manifestement à détourner le mécanisme de plafonnement des taxes affectées, dès lors que le dispositif comportait par ailleurs la possibilité de moduler à la baisse le taux de la contribution légale des acteurs concernés. Surtout, ce mécanisme paraissait incompatible avec le statut d'autorité publique indépendante de l'AMF,

un délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales, flanqué d'une délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, ainsi qu'une mission opérationnelle transfrontalière chargée de conduire trois missions, dans un dialogue avec les autorités nationales et européennes. Vous trouvez également beaucoup de moyens dispersés dans des cofinancements multiples, dont un programme appelé « NUTS »- ça ne s'invente pas ... Vous trouvez en outre des programmes de coopération territoriale- France-Espagne-Andorre, France-Belgique, Deux Mers, Rhin supérieur, France-Angleterre, Grande Région, Espace alpin, Espace atlantique, Espace méditerranéen -, ainsi qu'un fonds d'urgence humanitaire, des politiques de développement, des instruments de coopération territoriale. tout cela s'ajoutent les outils de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et du Conseil des communes et régions d'Europe. Tous travaillent « sur l'assistance de nos entreprises » à l'exportation.

et pour les territoires particulièrement touchés par la désindustrialisation. Dans le projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a décidé de diviser par deux le montant réservé au FDES. Alors que la situation économique de nos entreprises est encore fragile, il ne semble ni raisonnable ni réaliste d'opérer cette importante diminution des fonds dédiés au FDES. Cet amendement vise donc à revaloriser les crédits de paiement du programme « Prêts pour le développement économique et social

des repreneurs viennent taper à la porte, il y a bien sûr la BPI et d'autres opérateurs, mais cela ne suffit pas. On en a l'exemple avec Ascoval. Vous avez des porteurs de projets qui, après avoir fait l'objet d'études

que, derrière, l'absence du FDES montre que le Gouvernement ne croit pas au projet, comment les banques viendront-elles ? Comme pour le FISAC, quand il manque un élément au dispositif, malheureusement, cela met en péril des projets

plus qu'urgent de maintenir ces crédits. On le voit, cette année, ils vont être consommés. Ils sont utiles ! Ils sont attendus ! S'ils manquent au tour de table dans un projet aussi significatif que celui dont nous parlons ou dans ceux qui ne manqueront pas d'arriver, nous aurons un vrai souci. En l'état actuel des choses

industrielle pour notre pays. Cette force et cette vocation, j'ai eu l'occasion de les voir en Île-de-France lorsque je présidais la commission des finances de la région. Parfois cela ne me plaisait guère, mais nous aidions des entreprises à se restructurer, à redémarrer, et nous avons eu

La mise en place de solutions de redressement repose sur la capacité des différentes parties prenantes, notamment l'État, à se positionner rapidement. C'est pour cette raison que l'article 85 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder des remises de créances de prêts contractés auprès du FDES